La séance est reprise. Madame la ministre, mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande, en application de l'article 48, alinéa 3, de la Constitution,

Acte est donné de cette demande. En conséquence, l'ordre du jour du lundi 25 juin 2018 s'établira comme suit :- Suite du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie.

du scrutin. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie.

Rappelons historiquement que, en 1993, Charles Pasqua a porté ce nombre maximal de jours de 7 à 10 ; que Nicolas Sarkozy l'a augmenté à 32 jours en 2003, avant que Brice Hortefeux ne parachève ce travail de durcissement inique de la rétention des étrangers en portant ce nombre à 45 en 2011. Dans la version initiale du texte, le ministre d'État, Gérard Collomb, accomplissait l'exploit outrancier de doubler la durée maximale de rétention, en la portant à 90 jours, et ce sans la moindre justification légitime.

a décidé, à raison, de maintenir le chiffre déjà bien trop élevé de 45 jours. Cet article reste malgré tout problématique, par les autres dispositions qu'il contient. notamment à la possibilité, pour les préfectures, de placer en rétention un étranger soumis au règlement de Dublin refusant de donner ses empreintes, les altérant volontairement ou dissimulant des éléments de son parcours migratoire, de sa situation familiale et de ses demandes antérieures d'asile. Mes chers collègues, la manière dont sont traités ceux que l'on appelle les « dublinés » n'est pas acceptable. Les demandeurs d'asile ne sont pas en situation irrégulière, ils exercent un droit fondamental que nous devons leur garantir. Les faire sans cesse passer pour des escrocs et des criminels ne fera pas oublier le manque de courage de ceux qui ne veulent réformer ni les accords du Touquet ni le règlement de Dublin. La

et les policiers qui doivent gérer ces problèmes essaient de trouver les moyens d'agir au mieux. Mais les policiers ne sont pas des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire. Ils le disent eux-mêmes : ce n'est pas leur travail

Selon les chiffres de la direction générale des étrangers en France publiés sur le site du ministère de l'intérieur, lesquels sont, il est vrai, peu actualisés, le taux de délivrance des laissez-passer consulaires est assez faible. En 2011, le taux de délivrance global était de 32 %, et le taux de délivrance dans les délais de 29,5 %. Or, toujours en 2011,

Sauf à ce que ces résultats aient sensiblement évolué, nous sommes donc opposés à l'allongement proposé, qui pourrait se révéler à la fois coûteux pour le contribuable et dommageable pour les personnes placées, puis relâchées, faute d'obtention de ce fameux laissez-passer.

En outre, l'état de santé physique et psychologique des personnes placées en CRA, lesquelles sont affectées par la privation de liberté, ne permet pas un placement si long. Dans ces conditions, ni la solution proposée par le Gouvernement ni celle proposée par le rapporteur ne sont tout à fait acceptables. de supprimer l'essentiel de cet article, pour en rester au droit en vigueur, à l'exception des dispositions introduites par l'Assemblée nationale visant à mieux protéger les personnes vulnérables placées en centre de rétention administrative.

irrégulière et doit garantir en même temps l'accès de l'étranger à un recours effectif. La directive Retour ne définit pas le délai dans lequel doit intervenir le contrôle juridictionnel de la rétention, toutefois, son article 15 requiert que ce contrôle intervienne « le plus rapidement possible à compter du début de la rétention ». Une telle exigence est, du reste, conforme au paragraphe 4 de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme, qui garantit à toute personne privée de sa liberté « le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. La validation constitutionnelle obtenue le 9 juin 2011 sur la loi du 16 juin 2011 qui a reporté l'accès aux juges à l'expiration du cinquième jour ne suffirait pas à justifier un retour à une phase administrative de 5 jours. Dans le dispositif issu de la loi de juin 2011, l'accès au juge des libertés et de la détention était reporté au cinquième jour à l'occasion de l'audience contradictoire sur la requête aux fins de prolongation de rétention. L'étranger ne disposait pas d'un accès effectif rapide devant un juge compétent pour contrôler à la fois la privation de liberté et la légalité de la décision administrative de placement. Considérant la possibilité d'exécution de l'éloignement avant que le juge judiciaire ait statué, la Cour européenne des droits de l'homme a ainsi jugé que ces dispositions issues de la loi de juin 2011 n'étaient pas conformes aux exigences de la convention. Dans cette décision, la Cour a cependant pris acte de la réforme intervenue en mars 2016 en ce qu'elle a ouvert un droit de recours à l'étranger devant le juge des libertés et de la détention, suivant la notification de la décision de placement.

Au regard de la restriction de liberté que constitue ce placement, il est proposé de maintenir ce délai à 48 heures, afin que les personnes susceptibles d'obtenir la suspension de leur rétention puissent le faire valoir le plus tôt possible.

et de la détention. De nombreuses associations, dont la CIMADE, ont dénoncé des expulsions dites « sauvages » par lesquelles l'étranger est reconduit à la frontière alors même que le juge n'a pas statué sur sa requête. Ainsi, le collectif « Stop Dublin-Marseille » a publié en janvier dernier quelques témoignages sur les conditions d'arrestations et d'expulsions de demandeurs

parfois même contre des décisions de justice : « absence de traductions et d'interprètes à toutes les étapes de la procédure d'expulsion, pressions policières et menaces pour obliger les demandeurs d'asile à signer des papiers dont ils ne comprennent pas le contenu, escortes policières surnuméraires et entraves- menottes, liens pieds et jambes -non conformes à la situation, décisions de la préfecture de maintenir des expulsions alors même que des juges ont ordonné la remise en liberté ... » Sous couvert du règlement de Dublin, les polices pourraient donc aujourd'hui faire abstraction des lois, des décisions juridiques et du droit d'asile, ce qu'aucun d'entre nous ici ne saurait cautionner. cet amendement, deux propositions. Premièrement, la personne en rétention ne pourrait être éloignée du territoire avant que le juge des libertés et de la détention ait statué. Deuxièmement, tout agent public ayant pris une décision d'éloignement du territoire alors que le recours devant le juge est suspensif serait passible de poursuites. De plus, tout agent public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de tels actes et s'étant abstenu volontairement soit d'y mettre fin, s'il en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, serait passible des mêmes

La motivation de cette augmentation était la nécessité d'obtenir plus de laissez-passer consulaires afin de pouvoir s'assurer d'un renvoi vers les pays sources des retenus.

probablement pas d'améliorer nettement le taux d'éloignement des étrangers placés en rétention. » Il recommandait donc de « maintenir la durée maximale de rétention à 32 jours ». C'était le débat à l'époque.

en référence à des types d'états de santé, de handicaps ou de troubles psychiques, mais procède bien d'une évaluation individuelle

et refusant de donner ses empreintes ou les altérant volontairement. Cette disposition revient à permettre le placement en rétention des personnes qui refusent de donner leurs empreintes digitales, sans aucune autre condition et de manière systématique, sur la simple suspicion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 d'une personne ayant dissimulé des éléments de son parcours migratoire, de sa situation familiale et de ses demandes antérieures d'asile. Le critère permettant le placement en rétention pour dissimulation d'éléments de son parcours migratoire migratoire ou de sa situation familiale est flou et inadapté à la situation des demandeurs d'asile qui ont pu subir des traumatismes durant leur parcours. Il paraît dès lors raisonnable de penser qu'ils ne se confieront pas facilement à l'administration sur ces éléments. Par ailleurs, la loi permet de prendre en compte de manière suffisamment large toutes les situations

Quel est l'avis du Gouvernement ? Bien que le Conseil constitutionnel ait validé l'ensemble des dispositions de la loi Warsmann, l'Assemblée nationale s'est prononcée contre le maintien de ces deux critères ajoutés par le Sénat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

Si la rétention est néfaste pour des personnes ne présentant pas initialement de handicap, songeons aux répercussions qu'elle peut avoir sur celles et ceux qui sont, d'ores et déjà, en situation de handicap. Tout d'abord, à quoi bon retenir dans des centres de rétention des personnes en situation de handicap moteur, cognitif ou psychique, alors que le risque de fuite est bien souvent très faible, pour ne pas dire inexistant ?

Il est vrai que retenir des personnes handicapées en CRA apparaît comme une mesure inadaptée,. Ces personnes doivent faire l'objet d'un traitement à part entière, avec des mesures curatives idoines. Par ailleurs, le personnel n'est pas nécessairement formé à ce public, qui nécessite une attention toute particulière, et les moyens ne sont pas suffisants pour garantir des conditions décentes d'accueil et de soins. Par parallélisme, Par parallélisme, rappelons que la France a déjà été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme pour traitements inhumains ou dégradants, notamment le 4 février 2016 et le 23 février 2012, en raison des conditions de détention d'une personne atteinte de troubles mentaux. Tentons de ne pas encourir à nouveau les mêmes condamnations.

difficile. Quel est l'avis de la commission sur ces sept amendements

Quel est l'avis du Gouvernement ?

à la demande de séjour qu'à répondre à un besoin réel qui n'a jamais été démontré.

dans la rédaction actuelle le risque est d'entraîner une prorogation de la rétention pour raisons de santé, ce qui est totalement contraire à la demande de la personne, et éventuellement à ses droits. Cet amendement je vous remercie amplement développée, je ne vais pas la résumer une nouvelle fois. Je voudrais simplement saluer le courage et la lucidité de notre commission qui souhaite ramener le délai à 45 jours et qui s'en explique avec des arguments qui sont tout à fait recevables.

Nous n'arrivons pas à obtenir de retours volontaires en France alors qu'en Allemagne, c'est la politique générale. Il y a bien quelque chose à changer dans notre manière d'aborder l'éloignement,

pour qui ces questions sont des matières à conviction forte, que je ne suis pas d'accord avec eux. Je pense que nous ne devons pas transformer nos juges des libertés et de la détention en bureaucrates devant systématiquement, tous les jours, écluser des dizaines de cas qu'ils ont à peine le temps d'examiner. Ayons un certain égard pour nos magistrats ! Ce dispositif n'est pas efficace pour les étrangers en centre de rétention, car il induit une forme de routine dans le travail du magistrat. Par ailleurs, il existe un autre dispositif beaucoup plus efficace dont vous vous abstenez de parler, et qui suppose, tout simplement, soit soit que le juge des libertés prenne l'initiative de contrôles inopinés, soit que l'étranger, parce qu'il rencontre un problème sérieux, saisisse

dans la journée. Cela ne serait pas respectueux du travail d'un magistrat, qui doit se porter sur les difficultés sérieuses et réelles qui lui sont soumises et non entrer dans une routine administrative. C'est la raison pour laquelle je crois que, pour la protection de l'étranger

c'est la fermeture hermétique des frontières et un flux zéro, nous ne pourrons pas avoir une politique nationale, française ou allemande, digne de ce nom.

l'amendement n° 71. Par cet amendement, nous proposons de revenir sur l'augmentation à 10 heures du délai pendant lequel une personne déjà libérée par le juge des libertés et de la détention peut rester à la disposition de la justice, dans l'attente de la décision du parquet. Cette durée de 10 heures pour convenance de l'administration est, à la fois, injustifiée et excessive, d'autant que ce délai a déjà fait l'objet l'objet d'un allongement en 2011. Il a été porté de 4 à 6 heures, au motif, déjà, d'accorder plus de temps au procureur de la République pour solliciter le président de la cour d'appel, afin qu'il suspende la levée de la rétention.

chers collègues, les conditions concrètes de vie dans les centres de rétention, les difficultés rencontrées par un certain nombre de personnes qui y sont retenues. Dès lors, il nous semble que, s'il est possible d'organiser une audience par vidéoconférence lorsqu'une personne présente un recours contre une décision de prolongation de maintien en rétention, il faudrait que cela fût avec l'accord de la personne.

qu'un étranger placé en rétention ne puisse plus s'opposer à un jugement par vidéo-audience devant le tribunal administratif chargé de se prononcer sur la mesure d'éloignement. Nous avons dit, tout au long des débats précédents, notre réticence à voir se développer la vidéo-audience de façon constante. Le droit à un procès équitable et le principe de publicité des débats se trouveraient amoindris par le développement de la vidéo-audience, qui fait prévaloir un impératif budgétaire et logistique sur le respect impératif des droits de la défense. C'est pourquoi, au travers de cet amendement, nous prévoyons de restaurer la possibilité, pour le requérant, de s'opposer à l'utilisation de la vidéo-audience.

La commission n'a pas changé d'avis : celui-ci reste défavorable.

L'attention particulière qui est due aux personnes en situation de handicap renvoie, bien sûr, l'administration au respect du principe de proportionnalité de la procédure

d'autant qu'au-delà de l'accueil des personnes placées en rétention, les services de l'État, les associations, les équipes sanitaires, ainsi que le public visiteur- famille, avocats -peuvent, eux-mêmes, se trouver en situation de handicap. C'est pourquoi il est proposé de substituer, à l'amendement adopté par les députés, une précision indiquant que le décret déterminera les conditions d'accessibilité adaptées aux lieux de rétention.

du centre de rétention et la saisine du médecin de l'OFII. À l'heure actuelle, un certain nombre de personnes gravement malades se voient

affirmait qu'au-delà d'une durée de 5 ans, le maintien de l'assignation à résidence des étrangers faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire devrait être justifié par des circonstances particulières. En conséquence, l'article 17 du présent projet de loi propose qu'au-delà d'une durée de 5 ans, la menace pour l'ordre public soit constitutive de circonstances particulières, permettant ainsi le maintien de l'assignation. Il est précisé que cette assignation pourrait être renouvelée tous les 5 ans, sans limitation dans le temps. S'il est sans aucun doute nécessaire de se questionner sur la constitutionnalité d'une disposition du droit français, l'interprétation qui est faite, ici, de la décision du 1 décembre 2017 me semble, à la fois, fallacieuse et erronée. En effet, en ne cherchant pas à encadrer vraiment le renouvellement des assignations à résidence, le texte permet, de fait, le renouvellement à perpétuité de ces mesures hautement attentatoires aux libertés individuelles. le ministre d'État, la privation de liberté à vie n'existe pas en France. En tentant de répondre à une inconstitutionnalité, vous en créez une autre

La désignation de plages horaires pouvant aller jusqu'à 10 heures, pendant lesquelles le migrant doit demeurer dans les locaux où il réside, paraît incompatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est notamment ce que défend l'UNICEF.

ailleurs, comme le relève l'Observatoire du droit à la santé des étrangers, de telles plages horaires risquent d'impacter fortement l'accès des personnes malades à leur suivi médical, d'autant plus lorsque l'infrastructure leur procurant les soins est éloignée de leur lieu de domicile. C'est pourquoi nous souhaitons exclure de l'assignation à résidence de longue durée, à la fois, les mineurs avec leurs familles et les personnes nécessitant un suivi médical journalier. Quel

l'amendement n° 126. Les avancées de ce projet de loi sont assez rares pour être notées. L'une d'elles était l'article 17 , introduit à l'Assemblée nationale par la rapporteur du texte, la députée Élise Fajgeles.

le texte qui nous est présenté aujourd'hui prévoit donc le maintien des dispositions de la loi Warsmann. Le présent amendement tend à rétablir l'article 17 du projet de loi, c'est-à-dire réduire de 6 à 4 jours la durée de validité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention permettant aux forces de l'ordre d'effectuer des visites au domicile des assignés à résidence. La

afin de permettre aux forces de l'ordre d'effectuer des visites domiciliaires dans le cadre des assignations à résidence. C'est une mesure utile, laissant plus de temps à nos services pour agir. Ces amendements ayant pour objet de supprimer le dispositif, l'avis est défavorable.

Quel est l'avis de la commission ?

à savoir l'allongement de la durée de la retenue administrative de seize Depuis 2012, à la suite d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, le droit européen interdit le recours aux gardes à vue pour les demandeurs d'asile.

En délicatesse avec les préconisations légales européennes, cette mesure va également à l'encontre de l'avis que le Conseil d'État a rendu sur ce projet de loi en février 2018. Celui-ci rappelait alors que les demandeurs d'asile ne doivent pas être regardés en tant que tels comme des personnes en situation irrégulière, leur présence sur le territoire étant justifiée

des demandeurs d'asile, alors même que ces derniers n'ont pas commis le moindre fait répréhensible au regard de la loi et du droit. Ces exilés, qui ont parcouru un trajet difficile pour arriver en France, afin d'échapper aux divers bouleversements qu'ils ont subis dans leurs pays d'origine, méritent un traitement plus digne.

de la garde à vue, puisqu'il y est indiqué que « ce régime est calqué sur celui de la garde à vue alors que les deux mesures répondent à des finalités différentes et donc placent l'intéressé dans une situation juridique sans comparaison ».

de la situation juridique de la personne étrangère. Bien entendu, cette situation n'était pas acceptable du point de vue du respect des droits les plus élémentaires de la personne humaine. Elle introduisait une véritable

Depuis une loi du 31 décembre 2012, une procédure dite de « retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour », quelles que soient les garanties apportées, entraîne des conséquences sanitaires en matière de restriction des libertés.

instaurée par la Constitution, en particulier la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui en fait partie intégrante, la personne étrangère

comme tous ceux qui se mobilisent aujourd'hui contre le renforcement de la pression sécuritaire à l'encontre des étrangers, est dans une tout autre logique que celle du Gouvernement et de la majorité sénatoriale. Ceux-ci épousent la pensée de plus en plus dominante, qui désigne l'étranger comme un bouc émissaire.

et créé, en lieu et place de la garde à vue, une retenue aux fins de vérification du droit de séjour. Considérant que la procédure de vérification d'identité prévue à l'article 78-3 du code de procédure pénale, laquelle ne peut excéder quatre heures, était insuffisante pour la vérification du droit de circulation et de séjour, le législateur a décidé de créer un régime privatif de liberté spécifiquement dédié aux étrangers, d'une durée maximale de seize heures- heures. Cette durée permettait d'assurer « un équilibre entre les droits de la personne retenue, tant au regard de la privation de liberté que de la défense de ses intérêts, et les exigences qui s'imposent à l'autorité administrative Partant du principe que ce délai est actuellement excessif, il est essentiel que, au-delà de quatre heures, durée maximale de la garde à vue, des explications

Or c'est précisément l'objet de la retenue pour vérification ! La présence de l'avocat doit, dès lors, être prévue dès la première audition, sans restriction. Ce serait logique ! Cet

qui vise à permettre aux forces de l'ordre de retenir un étranger le temps de contrôler son identité. Le droit en vigueur prévoit que cette retenue ne peut être prolongée au-delà de seize heures, une durée déjà jugée excessive. Nous rappelons que l'Union syndicale des magistrats suggère, de façon constante, une réduction de ce délai maximal. L'alinéa 6 de l'article 19 prévoit au contraire d'étendre cette durée à vingt-quatre heures, en plus de la possibilité de collecter des empreintes digitales et des photographies, qui seront dans certains cas mémorisées. S'il peut être légitime de développer des moyens destinés à faciliter l'identification des personnes retenues, l'allongement de la durée de retenue est en revanche excessif. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cette disposition.

Tous ces amendements, sans exception, visent à remettre en cause, soit la totalité, soit certains aspects du régime de retenue pour vérification du droit de séjour. droit de séjour. Je rappelle que les diverses modifications procédurales proposées répondent à des besoins opérationnels : elles facilitent la lutte contre certains comportements d'obstruction ; elles permettent d'établir plus facilement la situation d'un étranger qui ne satisfait pas à l'obligation qui lui est faite de présenter les documents l'autorisant à circuler ou à séjourner en France ; enfin, elles permettent d'en tirer les conséquences s'il apparaît

Nous discutons d'une loi sur l'immigration et l'intégration : le fait de travailler en France, d'avoir un contrat de travail, de payer des droits sociaux n'est-il pas déjà

Or le CESEDA prévoit un contrôle des documents en vertu desquels les personnes de nationalité étrangère sont autorisées à circuler ou à séjourner en France. Ainsi, en fonction des circonstances dans lesquelles le contrôle est effectué, si l'intention manifeste de la personne contrôlée n'est pas de séjourner sur le territoire, l'incrimination prévue à l'article 441-8 du code pénal pourrait ne pas être mise en oeuvre. Ces situations se manifestent avec une particulière acuité à Mayotte. L'ajout du verbe « circuler » à l'article 441-8 du code pénal est justifié par la nécessité d'assurer la concordance entre les faits incriminés et leur qualification pénale.

amendement vise à retirer de la liste des autorités et personnes privées devant transmettre au préfet les documents et informations nécessaires à ses missions de contrôle les établissements scolaires et d'enseignement supérieur, les fournisseurs d'énergie et services de communications électroniques et les établissements de santé. En effet, la transmission de ces données porte une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée. ce dispositif n'est assorti d'aucune sanction en cas de non-réponse par les organismes visés. De ce fait, il engendre une inégalité entre les personnes contrôlées, selon que les établissements répondent ou non aux demandes formulées par l'autorité administrative.

si un placement dans un centre de rétention administrative a été demandé. Or, au regard des taux élevés d'inexécution des décisions d'OQTF, il est indispensable d'élargir cette possibilité de sanction pénale à toute inexécution d'OQTF, avec ou sans placement en centre de rétention administrative, ainsi qu'à toute inexécution d'interdiction du territoire français judiciaire ou d'assignation.

en cas de placement en rétention, n'a pas vu expirer la durée maximale de celle-ci. Ce dispositif n'interdit heureusement pas aux législateurs nationaux de sanctionner pénalement le maintien sur le territoire en dépit d'une mesure d'éloignement, ainsi que le fait de se soustraire à l'exécution d'une

avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. L'article 19 A prévoit des sanctions en cas de méconnaissance par un étranger d'une mesure d'éloignement. Pourtant, la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour de cassation ont jugé qu'on ne peut appliquer une mesure d'emprisonnement à un étranger s'il peut encore être recouru à son égard à la rétention. La directive Retour prévoit en effet que la procédure administrative, c'est-à-dire la rétention, ne peut pas être entravée par une peine d'emprisonnement. L'article n'est pas conforme à cette jurisprudence, puisque, dans de nombreux cas, la peine d'emprisonnement serait possible quand bien même il pourrait encore être recouru à la rétention.

Toutefois, en l'espèce, il convient de ne pas surinterpréter la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne sur les exigences résultant de la directive. Celle-ci doit être comprise comme tendant à favoriser la mise en oeuvre des mesures d'éloignement, non à l'entraver. Ainsi, lorsque c'est l'obstruction de l'étranger lui-même qui s'oppose à l'exécution de la mesure d'éloignement, par exemple sous la forme d'un refus d'embarquement, son comportement justifie la mise en oeuvre d'une procédure judiciaire. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît l'effet utile de sanctions pénales, y compris d'emprisonnement, lorsqu'elles contribuent par leur effet dissuasif à la réalisation des objectifs de la directive Retour.

Darcos. Je présente cet amendement au nom de notre collègue Brisson. Donner à l'autorité judiciaire la possibilité de prononcer une interdiction judiciaire du territoire français pour tout délit puni d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois permettrait d'inclure les infractions telles que le vol, le vol avec violences avec une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, le recel, l'escroquerie, l'abus de confiance, la contrebande, le travail clandestin, les menaces de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique, les violences aggravées

L'objectif est d'offrir à nos forces de sécurité intérieure une liberté plus grande, afin de lutter efficacement contre l'immigration clandestine, qui va vraisemblablement s'intensifier, puisque l'Italie ne reprendra plus ses clandestins. La police aux frontières, que le Gouvernement vient de renforcer préventivement, va vivre des moments difficiles

Par ailleurs, l'amendement tend à donner la possibilité aux officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, aux agents de police judiciaire de procéder à des fouilles de bagages et à des visites de véhicules au sein des départements frontaliers, dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière.

l'accompagnement linguistique et social de l'étranger, ainsi que tout transport lié à l'une de ces exceptions, sauf si l'acte a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte ou a été accompli dans un but lucratif.

Avec le dispositif que nous proposons, passeurs et solidaires ne seront plus confondus. La preuve de la culpabilité sera désormais à la charge de l'administration, et non plus de ceux qui sont aujourd'hui criminalisés pour leurs actions humanitaires. Il n'est pas normal que des Justes du XXI siècle, traités de délinquants solidaires, comme Pierre-Alain Mannoni, Cédric Herrou, Martine Landry et d'autres, encourent

migrants. En dépit des modifications successives apportées par le législateur, la pénalisation des actions menées par des citoyens à l'égard des migrants dans la détresse demeure. De fait, la pénalisation de l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers a été déviée de sa cible. Elle devait avoir pour objectif de poursuivre et sanctionner les personnes et organisations qui font avec les réfugiés un trafic humain lucratif, exploitant la misère et maintenant dans un état de dépendance les personnes qui souhaitent entrer sur le territoire français pour faire valoir leur droit à l'asile. Les modifications apportées au dispositif par l'Assemblée nationale ne sont qu'une rustine, qui n'empêchera aucunement les humanitaires, bénévoles et citoyens d'être poursuivis et, le cas échéant, condamnés, alors même qu'ils ont agi sans contrepartie et guidés par le seul désir de porter secours à des hommes, des femmes et des enfants. Le mécanisme d'exemption prévu à l'article L. 622-4 est complexe et ambigu. Il fait régulièrement la preuve de son inefficacité, en faisant condamner des citoyens qui, de toute évidence, ne sont pas des passeurs. Il faut donc changer de logique : rompre avec une logique d'exemptions et redéfinir globalement l'incrimination d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers. Tel est l'objet de cet amendement, qui intègre deux éléments constitutifs pour qualifier l'infraction. D'une part, le caractère intentionnel de l'acte : il devra être prouvé que les intéressés ont agi dans l'intention de commettre l'infraction. D'autre part, le caractère lucratif, car les actions menées à titre gratuit, sans recherche de profit, signifient qu'elles poursuivent une ambition humanitaire et ne peuvent donc être poursuivies. En vertu de la rédaction que nous proposons, les passeurs qui agissent avec l'intention de commettre une infraction et dans un objectif de profit continueront à être poursuivis et condamnés. À leur égard, l'État ne doit faire preuve d'aucune indulgence. Cet amendement ne fait preuve d'aucune indulgence à leur endroit. En revanche, nous redéfinissons le cadre, de manière à abroger

à M. Maurice Antiste. Depuis 2014, les poursuites et condamnations contre des citoyennes et citoyens solidaires avec les personnes étrangères se sont multipliées en France, y révélant la persistance du délit de solidarité. Alors qu'il était prévu que l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permette de pénaliser les personnes et les organisations qui font du passage illégal des frontières un hautement lucratif, force est de constater aujourd'hui qu'il sert toujours à poursuivre, voire à condamner, celles et ceux qui, par solidarité, refusent de laisser sur le bord de la route des personnes étrangères démunies. En 2012, la loi Valls promettait la fin de ce délit de solidarité avec l'extension des critères d'immunité. Dans les faits, les poursuites et les condamnations de citoyens et de citoyennes solidaires se sont multipliées, par exemple dans le Calaisis, à Paris, dans la vallée de la Roya, à Briançon et ailleurs. C'est pourquoi ma proposition prend en considération les contraintes découlant de la directive du 28 novembre 2002, qui oblige les États membres à pénaliser l'aide à l'entrée, au transit et au séjour, sauf but humanitaire ou absence de but lucratif, en maintenant cette qualification spécifique, mais en délimitant beaucoup plus nettement son champ d'application. Plus précisément, il s'agit d'exclure du champ des poursuites, de manière véritablement explicite, les actions purement désintéressées ou qui relèvent de la fourniture normale d'un bien ou d'un service. De plus, le mécanisme de l'immunité institué à l'article L. 622-4, complexe et ambigu, ayant démontré son inefficacité, la définition de l'infraction serait modifiée, à travers notamment la suppression de la notion d'aide, la notion de circulation, l'interdiction de territoire français et le remplacement de la mention directe ou indirecte » par le terme « sciemment », figurant dans la directive. Cet amendement répond donc à l'objet de la directive et permet de redonner tout son sens à l'infraction pénale, qui vise à lutter contre les réseaux de passeurs et l'exploitation subie par les personnes migrantes, tout en excluant de son champ les actes de solidarité à l'égard des personnes étrangères en situation irrégulière.

éventuellement, idéologiques, pensent qu'on doit abolir les frontières et agissent pour que des gens puissent entrer en France de manière illégale, il n'est évidemment pas question pour nous de les laisser faire et de ne pas les sanctionner.

Leur action se substitue dans bien des cas à celle de l'État. L'engagement de certains d'entre eux les conduit parfois à vouloir faire changer les lignes de la politique d'accueil et pallier les limites du système non coopératif de Dublin.

Dans la perspective d'aider les aidants, la modification de l'article L. 622-4 du CESEDA adoptée par l'Assemblée nationale nous paraît avoir atteint un équilibre acceptable. C'est pourquoi nous proposons de la rétablir.

note qu'il y a d'abord un problème d'emploi des mots : il ne s'agit pas du délit de solidarité, mais du délit d'aide au séjour irrégulier sur le territoire national.

Dieu sait s'ils sont nombreux -, mais aussi, grâce au discernement des procureurs, de ne pas poursuivre ceux qui, de façon spontanée, généreuse, sans arrière-pensée de réseau à construire ou de bénéfice à retirer, apportent, à un moment ou à un autre, un soutien à un étranger en situation irrégulière. Ce que chacun d'entre nous serait tout à fait capable de faire- et ferait d'ailleurs sans aucun doute.

L'état des forces en présence est clair : la gauche souhaite une réelle abrogation du délit de solidarité ; la droite opte pour le maintien du droit existant, et l'exécutif, soutenu par la majorité présidentielle et le RDSE, nous propose une révision en trompe-l'oeil du délit de solidarité. Avant que, toutes et tous, nous nous prononcions en votant sur les différents amendements qui nous sont soumis, il me semble important de vous rappeler, mes chers collègues, qu'il ne s'agit pas ici de polémiquer sur les orientations de la politique migratoire. Il s'agit de montrer le véritable harcèlement dont sont victimes des femmes et des hommes qui font preuve d'humanité envers leurs semblables et d'y mettre un terme. Ce n'est pas la première fois que, devant l'émotion provoquée par les vagues de poursuites et de condamnations de personnes solidaires, le ministre de l'intérieur en poste prétende abroger cette incrimination indigne. tous ont annoncé, depuis vingt ans, la fin du délit de solidarité. Il n'en a rien été, et nombreux sont ceux qui pourraient en témoigner aujourd'hui. Ces solidaires, ces aidants, je les ai rencontrés partout en France, et ils sont loin de la caricature que certains veulent bien en faire. Ils sont retraités, infirmières, professeurs ou agriculteurs ; ils ont des valeurs humanistes avant tout, qu'ils soient de gauche ou de droite, et considèrent qu'un migrant est avant tout un être humain. Vous ne ferez pas exception, monsieur le ministre d'État, le dispositif que vous nous proposez est voué à produire les mêmes effets que les précédents prétendus assouplissements. Aussi, je vous demande, mes chers collègues, quelles que soient vos convictions en matière d'accueil des exilés, d'envoyer un message fort à nos concitoyens, un message de solidarité et de fraternité en adoptant l'amendement que je propose avec mon groupe. Pour finir, je tiens à vous dire, monsieur le rapporteur, que vous avez de nouveau fait, probablement exprès, la confusion entre passeurs et solidaires.

explication de vote. Les mots ont un sens. Lorsqu'on parle de nouveaux Justes, de qui se moque-t-on ? Les Justes, pendant la guerre- faut-il le rappeler ici ? -, risquaient leur vie pour aider les juifs ou ceux qui étaient persécutés par les nazis. Employer ces termes aujourd'hui dans cet hémicycle est complètement indigne. Que risquent-ils maintenant ? D'aller à Cannes

Mes chers collègues, on ne peut pas continuer à confondre le bénéfice, l'enrichissement personnel de quelques-uns, que nous dénonçons tous, avec un acte militant,

on assiste à des débats extrêmement inquiétants. On ne peut considérer comme vous le faites, mon cher collègue Bascher, que l'assistance à personne en danger peut être invoquée, parce que, malheureusement, bien souvent, personne n'est là

de gens qui accompagnent sans relation vénale, sans relation de domination, sans relation d'aliénation et sans relation d'exploitation. Je pense

Nous sommes en France, et c'est une démocratie. Nous sommes en France, et nous votons. Nous sommes en France, et il y a un parlement, un gouvernement, des lois. Et ces lois-

Pour notre part, ni explicitement ni implicitement, nous ne l'avons fait. Ensuite, je reprendrai les propos de Roger Karoutchi lui-même : notre pays est une démocratie, et nous sommes au Parlement. Nous estimons que la discussion parlementaire d'aujourd'hui est l'occasion de proposer et, espérons-le, d'adopter la suppression du délit de solidarité.

est sexiste ! Madame Benbassa, nous ne sommes pas là pour émettre des messages forts ou des signaux faibles, mais pour faire la loi.

Je me permets de vous signaler, et j'espère ne pas vous mettre en colère, que le délit de solidarité n'existe pas dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Effectivement ! Je suppose que, s'il avait existé, la loi du 31 décembre 2012 proposée par le gouvernement de M. Ayrault l'aurait immédiatement supprimé. Il ne l'a pas fait, et vous ne vous en êtes pas plainte à cette époque, me semble-t-il, mais peut-être corrigerez-vous cette appréciation si elle se révèle inexacte.

contre une nouvelle forme de traite que constitue le trafic des passeurs, qui font entrer clandestinement, en France et dans d'autres pays d'Europe, des étrangers généralement démunis et vulnérables. C'est donc une assistance aux étrangers eux-mêmes

la mise en cause de Français agissant soit en raison de liens familiaux, soit par pur désintéressement et sens de la fraternité. De ce point de vue, on peut partager votre motivation, à condition qu'elle s'appuie sur la réalité du droit. Or j'ai tenté d'expliquer que le droit n'est pas tel que vous l'avez décrit. La loi du 31 décembre 2012

cette personne peut être poursuivie pour un délit. C'est bien naturel, parce que cette contrepartie atteste qu'il ne s'agit pas d'un acte de fraternité. Mais, s'il n'y a pas de contrepartie, les les poursuites n'ont pas lieu d'être. Si, par erreur, il y avait quand même des poursuites, le tribunal ne pourrait pas condamner, sinon cette condamnation serait naturellement annulée en appel. Je trouve que la loi n'est pas si mal faite. faite. Elle prend en considération les préoccupations que vous exprimez. Je pense, par conséquent, qu'il faut la maintenir dans ses grandes lignes, sans lui donner de coups de boutoir, ce qui reviendrait à à inciter les passeurs à développer leur coupable commerce au détriment de malheureux qui franchissent les océans au péril de leur vie pour rejoindre l'Europe.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

le même temps, nous constatons que d'autres personnes, souvent animées par des idéologies racistes et xénophobes, participent, en toute impunité, à des actions scandaleuses destinées à entraver l'exercice du droit d'asile. Il apparaît particulièrement inadmissible que de telles actions, parfois d'une extrême violence psychologique ou physique, puissent perdurer sans que leurs auteurs soient inquiétés. Malheureusement, des exemples récents démontrent que les étrangers sont fréquemment victimes de tels actes malveillants. Ainsi, des personnes physiques ou des groupuscules extrémistes constitués en association montent des opérations visant à empêcher des personnes étrangères d'entrer en France et d'y solliciter l'asile, postant des kilomètres de barrières à la frontière franco-italienne à renfort d'hélicoptères. D'autres leur communiquent de fausses informations ou les empêchent de se rendre auprès des autorités compétentes en vue de déposer une demande d'asile. Ils font tout cela sans être poursuivis et se vantent pourtant de leurs odieux actes sur les réseaux sociaux.

Un certain nombre de gens commettent des actes répréhensibles, d'un côté ou d'un autre, au nom d'idéologies souvent opposées. Nous n'accepterons pas que cela se perpétue, et toutes les personnes qui commettront des actions violentes seront poursuivies.

des actes particulièrement insupportables. Je profite donc de cette occasion pour défendre une conviction républicaine : le parquet doit rester à la disposition du Gouvernement au nom de l'action publique.

Dans son avis relatif à l'évaluation de la minorité d'un jeune étranger isolé, rendu le 23 janvier 2014, le Haut Conseil de la santé publique a notamment indiqué qu'avec la méthode couramment employée, reposant sur une radiographie de la main et du poignet gauche du jeune, laquelle est comparée avec des clichés de référence,

médecine et les décisions et les propositions du Défenseur des droits, nous proposons une interdiction complète des tests osseux.

vous l'a dit, aujourd'hui, les processus physiologiques font que certains grandissent mieux et plus vite que d'autres. J'en suis un peu le témoignage vivant.

Il faut donc pouvoir repérer les enfants mineurs de façon quasi certaine, tout en évitant l'instrumentalisation des dispositifs. La commission des lois souhaite s'appuyer fortement sur la loi de 2016 relative à la protection de l'enfance, qui

Les examens radiologiques osseux visant à déterminer l'âge ne peuvent être réalisés qu'en second lieu. Ils sont entourés, évidemment, de plusieurs garanties : ils ne sont réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire, après recueil de l'accord de l'intéressé ; les conclusions de ces examens doivent préciser la marge d'erreur et ne peuvent, à eux seuls, permettre de déterminer si l'intéressé est mineur, et le doute lui profite toujours.

Madame la présidente, monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, je veux dire à Mme Benbassa que, si je me suis emporté tout à l'heure- le président de la commission a parlé de « sainte colère » -, ce n'est pas trop mon habitude. Je déteste me mettre en colère dans l'hémicycle. Je lui présente donc mes excuses

Mes collègues socialistes membres de la commission de la culture et moi-même nous sommes particulièrement intéressés aux articles 20 à 22 de ce projet de loi, car ils concernent le séjour et l'accueil des « talents », c'est-à-dire les chercheurs, créateurs d'entreprise, investisseurs, ceux qui exercent des emplois qualifiés ou des activités sportives ou artistiques, mais aussi le séjour des étudiants et chercheurs qui suivent un programme de mobilité, sans oublier des jeunes au pair. L'article 20 vise à élargir les critères de délivrance du « passeport talent », que le Gouvernement précédent avait prévu dans la loi du 7 mars 2016. Reconnaissant le succès du dispositif, le projet de loi prévoit, par exemple, d'étendre la possibilité de délivrance d'un « passeport talent » aux salariés de toutes les entreprises innovantes et non plus seulement aux salariés des jeunes entreprises innovantes. Il est également prévu une extension du « passeport talent » à tous les enfants du couple, ce qui permet de reconnaître les familles recomposées. Transposant la directive du 11 mai 2016 dite « Étudiants-chercheurs », l'article 21 prévoit la création de cartes de séjour pour les étudiants et chercheurs relevant d'un programme de mobilité comme Erasmus Mundus ou Marie-Curie. Il est également prévu de faciliter leur séjour lorsque, à l'issue de leurs études ou recherches, ils souhaitent créer une entreprise ou cherchent un emploi en France. L'article 22 résultant également de la transposition de la directive de 2016 prévoit un statut pour les jeunes au pair, qui, jusqu'à maintenant, se voyaient délivrer une carte de séjour « étudiant ». Même si ces mesures étaient inéluctables, puisque résultant d'une directive européenne, Mme Lepage se réjouit des dispositions favorables qui ont été introduites. qui ont été introduites. Elle se réjouit également du choix du Gouvernement de suivre la droite ligne de l'action du gouvernement précédent en ce qui concerne l'accueil des « talents ». Cela lui permet d'affirmer que ce qui est prévu dans les articles 20 à 22 de ce projet de loi va dans le bon sens, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble de ce texte.

Cet amendement vise à ajouter les projets culturels, sportifs, sociaux ou scientifiques. En réalité, il est déjà satisfait par un autre critère de délivrance du « passeport talent », qui concerne les projets dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif, artisanal ou sportif.

Quel est l'avis de la commission ?

vise à insister sur la nécessité de développer davantage d'outils de codéveloppement entre les pays d'origine et les pays de destination des migrations internationales actuelles. La formation d'élites économiques aux métiers d'avenir ou aux activités nécessaires au développement soutenable des pays d'origine pourrait recevoir un meilleur accompagnement sous la houlette de l'Agence française de développement. Le développement de relations d'un nouveau type avec les ressortissants des pays d'origine pourrait être un instrument efficace du rayonnement français à travers le monde. Tel est l'objet de cet amendement.

quelques éléments, sans vous abreuver de statistiques. Je prendrai simplement l'exemple d'un pays du Maghreb, la Tunisie. Depuis très longtemps, la majorité des étudiants tunisiens viennent étudier en France.

pour des cursus en anglais. Je pense que cela ne sert ni notre pays ni la francophonie. Je voudrais vous citer un autre exemple, celui du Cameroun. Le nombre d'étudiants camerounais qui viennent étudier en France a baissé de près de 25 %, au

laquelle se soumettent bien volontiers les étudiants français. Si nous n'arrivons pas à offrir des capacités d'accueil aux étudiants étrangers, ils iront

un accord de l'espace Campus France, quelqu'un se rend au consulat pour demander son visa étudiant, il ne peut savoir si l'espace Campus France a donné un avis favorable ou défavorable à son projet.

par la commission, fusionne de façon malencontreuse les cartes de séjour temporaires et les cartes de séjour pluriannuelles. Or ces deux titres ne répondent pas aux mêmes objectifs et ne s'appuient pas sur les mêmes critères.

aboutir à un dispositif un peu plus lisible en créant des articles spécifiquement dédiés à la mobilité européenne des étudiants étrangers. Le titre mixte ainsi créé s'inspire, par exemple, du titre de séjour des travailleurs en CDD, et il permettra des contrôles effectifs. D'autre part, la commission a souhaité que l'étudiant mobile justifie d'une connaissance suffisante de la langue de son programme d'études et d'une assurance maladie, comme le permet d'ailleurs la directive du 11 mai 2016.

S'agissant de celui que nous avons déposé et qu'a défendu mon collègue Pierre Ouzoulias, je voudrais vous rappeler, mes chers

qui est contre

nous propose, avec l'ensemble de notre groupe, d'adopter cet amendement qui a pour objet les étudiants étrangers, mais aussi les chercheurs. Aujourd'hui, les étudiants étrangers titulaires d'un diplôme de niveau bac+5, d'un doctorat ou d'une licence professionnelle peuvent se voir délivrer une autorisation de séjour d'un an non renouvelable à des fins de recherche d'emploi salarié ou de création d'entreprise. Les chercheurs ne peuvent bénéficier d'une telle autorisation et doivent donc changer de statut pour obtenir un titre de séjour en qualité de créateur d'entreprise ou de salarié. La directive européenne Étudiants-chercheurs du 11 mai 2016 impose la création d'un titre de séjour spécifique pour permettre aux étudiants et aux chercheurs de rester sur le territoire national à des fins de recherche d'emploi ou de création d'entreprise. Le choix du Gouvernement pour appliquer cette directive a malheureusement été de créer une seule carte de séjour d'un an, non renouvelable, pour la création d'entreprise comme pour la recherche d'emploi. Or ces deux activités sont bien différentes et nécessitent un traitement distinct. En effet, la création d'une entreprise requiert souvent bien plus d'une année. Cet amendement vise donc à prévoir une distinction des deux situations et une possibilité de renouvellement de la carte de séjour en cas de création d'entreprise. L'amendement n° 391 rectifié, présenté par MM.

de revenir dans un délai de quatre ans pour y constituer son entreprise. Notre principe est que, une fois ses études terminées, il peut créer son entreprise sur le territoire, mais immédiatement.

permettre de renouveler ce titre de séjour lorsque l'étudiant ou le chercheur souhaite créer une entreprise. L'avis de la commission est défavorable, parce que ce titre de séjour est par définition de courte durée. Dès que le projet de création d'entreprise est plus avancé, l'étranger peut évidemment

partie intégrante du cursus. L'attractivité de la France en matière d'enseignement supérieur ne peut donc pas être séparée de la manière dont elle traitera

pour avis. Dans le droit en vigueur, la responsabilité du « suivi sanitaire préventif » des étudiants étrangers est confiée aux établissements d'enseignement supérieur. Auparavant, en vertu d'une disposition de nature réglementaire, les étrangers, étudiants comme non étudiants, devaient obligatoirement, pour valider leur visa, passer une visite médicale à l'Office l'OFII a fait passer 210 000 visites médicales, dont 60 000 concernaient des étudiants étrangers. Or ledit office, pressé par le Gouvernement de stabiliser ses moyens, souhaitait être déchargé de cette mission pour certaines catégories d'étrangers,

hors Union européenne présents dans les hôpitaux ne rempliront plus les conditions légales pour poursuivre leurs fonctions dans l'attente de l'obtention de l'autorisation d'exercer pleinement leur profession et de leur pleine intégration au système de santé français. Ils devraient de ce fait cesser leurs fonctions. s'agit donc de prévoir la coordination nécessaire au maintien d'un dispositif essentiel au bon fonctionnement de nos hôpitaux, notamment ceux pour lesquels le recrutement de praticiens médicaux se révèle difficile.

Cette dépendance est d'autant plus forte que le jeune en question se trouve dans un pays étranger, où il a logiquement peu de réseaux et peu de relais en cas de problème.

À ce titre, l'enquête de France Info publiée au mois de mars dernier et mise à jour au mois de mai est édifiante. On peut aussi rappeler que des enquêtes ont été menées dans plusieurs arrondissements parisiens et ont montré de graves abus, et ont montré de graves abus, au point qu'un certain nombre de députés du groupe Les Républicains de l'Assemblée nationale ont voté l'amendement identique proposé par ma collègue Marie-George Buffet,

La plupart des cas observés sont légalement répréhensibles. Encore faut-il que les jeunes soient en position d'engager des poursuites et se trouvent accompagnés. C'est la raison pour laquelle nous reprenons une préconisation du Comité contre l'esclavage moderne, en incluant dans la convention une annexe avec les coordonnées

présenter l'amendement n° 18. L'article 23 dispose qu'un étranger qui a déposé une demande d'asile et qui souhaite solliciter par ailleurs un titre de séjour pour un autre motif doit effectuer cette seconde démarche parallèlement à sa demande d'asile. Selon l'association d'avocats du droit d'asile ELENA, ce droit existe déjà, même si, en pratique, nombre de guichets refusent illégalement d'enregistrer ces doubles demandes

dublinés » n'auraient pas à être informés de ce droit dont ils disposent pourtant aujourd'hui, et le dépôt de la demande de titre de séjour serait encadré dans un délai qui serait fixé ultérieurement par décret en Conseil d'État.

Cela peut concerner la demande de réexamen, la découverte d'une pathologie, un changement de situation ouvrant de nouvelles possibilités de solliciter un titre de séjour. Toutefois, cette notion nous paraît particulièrement floue et nécessiterait d'être concrètement définie. Une nouvelle fois, il s'agit d'être rigoureux lorsqu'il y va du sort de femmes et d'hommes dont l'avenir est suspendu à une décision de l'administration. En outre,

Même avis. L'article 23 consacre explicitement le droit pour tout étranger demandeur d'asile de solliciter parallèlement son admission au séjour pour un autre motif. Par conséquent, le demandeur disposera d'une information- ce qui n'est pas le cas actuellement -et d'un délai suffisant pour déposer son dossier. En revanche, au-delà de ce délai, il ne pourra plus, sauf circonstances nouvelles, déposer de nouvelles demandes. Cet article constitue donc un réel progrès pour le demandeur, qui verra sa situation examinée de manière globale, dans un délai déterminé. Il permet de faciliter le travail de l'administration. Enfin, il contribue à améliorer la lutte contre des demandes dilatoires.

ne pourrait plus le faire, puisqu'elle ne l'aurait pas fait en même temps que sa demande d'asile. Elle se trouverait paradoxalement dans une situation que l'on pourrait qualifier de « ni-ni

Cet amendement vise à supprimer la restriction de circulation concernant les mineurs étrangers admis au séjour à Mayotte. Actuellement, le document de circulation pour étranger mineur, le DCEM, permet la réadmission du mineur sur l'ensemble du territoire français. L'article 24 prévoit désormais que les DCEM délivrés par le préfet de Mayotte ne permettront une ne permettront une réadmission de leur titulaire que sur le territoire de Mayotte. Ce régime dérogatoire viendra accentuer la pression sur un territoire qui ne parvient déjà plus à gérer le défi migratoire.

la prolifération de bidonvilles, la saturation des services publics de la santé, de l'éducation nationale, des réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement ou encore la dégradation accélérée de l'environnement et du lagon. C'est l'ensemble des politiques publiques de rattrapage du territoire le plus pauvre de France qui est mis en échec par l'augmentation de la démographie induite par l'immigration. Il est donc proposé que les titres de séjour délivrés par l'État à Mayotte permettent l'accès à l'ensemble du territoire. La

Je ne partage pas ses convictions, et il le sait, mais je pense qu'un sujet aussi important que le statut de Mayotte et la possibilité que cette île ne soit pas un territoire de droit commun associé à la République méritaient une petite réponse. pas un discours ni une leçon d'agrégation, mais une prise de position qui nous aurait permis de comprendre ce que le Gouvernement souhaite engager

La condition selon laquelle le mineur ne peut se voir délivrer un DCEM que s'il est né en France, lorsque l'un de ses parents est titulaire d'un titre de séjour, est justifiée par la situation particulière de Mayotte. C'est la raison pour laquelle l'avis de la commission est défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? ? Même avis que le rapporteur. L'article 24 prévoit que seuls les mineurs étrangers nés à Mayotte peuvent, lorsqu'ils y résident habituellement avec leurs parents, dont l'un au moins est en séjour régulier, prétendre à la délivrance de plein droit d'un DCEM, la condition relative à la naissance en France étant notamment de nature à garantir une meilleure authentification des actes d'état civil. Les mineurs nés à l'étranger qui résident habituellement à Mayotte peuvent néanmoins se voir délivrer un DCEM. En ce cas, la seule condition tenant au séjour régulier de leurs parents ne peut suffire : ces mineurs doivent également justifier d'une entrée régulière sur le sol français et être entrés avant l'âge de treize ans. La présentation d'un passeport revêtu d'un visa

aux mineurs qui ont vocation à obtenir un titre de séjour à la majorité. Aussi, à Mayotte, le mineur ne doit pas nécessairement être né en France pour pouvoir bénéficier de la délivrance d'un DCEM. S'il est né à l'étranger, il devra remplir des conditions supplémentaires, notamment celle de l'entrée en France sous couvert d'un visa. Cette mesure dérogatoire participe pleinement à la maîtrise des flux migratoires dans le contexte spécifique de Mayotte, où le détournement des dispositifs légaux peut conduire à l'instrumentalisation d'enfants à des fins migratoires et de fraude à l'état civil. J'ai essayé de vous faire la réponse la plus complète possible.

discours qu'il a prononcé l'été dernier à Orléans, le Président de la République a insisté sur le rôle essentiel que jouent la culture et l'éducation dans l'intégration des primo-arrivants. Naturellement, l'apprentissage de la langue et la connaissance des valeurs de la République, qui impliquent de faire un détour par l'histoire de France, sont fondamentaux. Néanmoins, l'intégration passe aussi par l'accès à la culture, l'éducation et le sport. Si l'éducation renvoie en partie à l'acquisition de savoirs, la culture et le sport suscitent un éveil de nature différente. En effet, la pratique culturelle et sportive fait entrer en jeu le lien social : alors que l'apprentissage de la langue ou des principes républicains peut se révéler solitaire, les activités culturelles et sportives se déroulent

Les interactions et échanges qui naissent sous ce jour favorisent le partage et l'intégration des primo-arrivants. Dans nos territoires, nous connaissons tous des associations culturelles ou sportives qui oeuvrent en ce sens. Nous savons leur importance pour l'intégration des primo-arrivants. N'oublions pas que, pour ces derniers, la pratique culturelle et sportive est parfois une échappatoire vitale à leur quotidien ou à l'expérience qui a précédé leur arrivée en France. En ce qui concerne plus spécifiquement la culture, sans faire de grand discours sur le sujet, je crois qu'il faut au moins rappeler à quel point il s'avère indispensable de la partager, afin d'intégrer dignement et réellement tous les facteurs de compréhension de notre pays et de ses habitants. C'est un vecteur d'intégration important. Jean Vilar, « la culture, ce n'est pas ce qui reste quand on a tout oublié, mais au contraire, ce qui reste à connaître quand on ne vous a rien enseigné. » Nombreux sont les exilés à qui beaucoup de choses ont été enseignées ; là ne réside pas la question. En revanche, cette idée que la culture est tout autant une conquête de l'espoir à s'approprier résonne profondément avec la vie des exilés à leur arrivée chez nous. C'est pourquoi il est proposé d'étendre les finalités du parcours d'intégration républicaine en prévoyant qu'il donne accès à la culture, à l'éducation et au sport dès le début.

et l'acquisition de la nationalité, qui sont normalement déterminés au niveau réglementaire, ont été introduits à l'article 26 B du projet de loi et ont été relevés par rapport à ceux qui sont actuellement demandés. Or ces derniers ont déjà été rehaussés récemment- en 2016 pour la carte de séjour pluriannuelle et en 2018 pour la carte de résident. Il n'est pas opportun d'augmenter encore ces niveaux.

En tout état, de cause, nous proposons de mettre en place, sur ce sujet, une transposition de la directive Accueil qui soit complète et conforme au droit européen. Aujourd'hui, nous ne sommes même pas en mesure d'établir

Ainsi, de nombreux réfugiés ou exilés se trouvent maintenus dans des conditions de dénuement qui nous semblent contraires à la dignité humaine et susceptibles de caractériser des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. Aussi, l'amendement que nous défendons vise à faciliter l'intégration des demandeurs d'asile en leur donnant la possibilité d'accéder à l'emploi six mois après l'introduction de leur demande. Je pense que

À la limite, le délai n'a pas beaucoup d'intérêt, si je puis me permettre cette expression : il faut l'apprécier en fonction du délai d'appréciation de la demande d'asile elle-même. Si nous sommes capables de traiter une demande d'asile

Il paraît très important de permettre à un étranger ayant fait des démarches en ce sens et n'ayant pas obtenu de réponse de l'administration dans un délai raisonnable d'accéder au marché du travail après six mois et non neuf. Nous le savons tous, le travail est un outil majeur pour favoriser l'intégration. L'amendement n° 136 rectifié,

n° 331 rectifié. Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 26 , supprimé par la commission des lois, concernant la délivrance de plein droit d'une autorisation de travail au mineur isolé étranger qui a été confié à l'ASE. proposée par le rapporteur, au motif que cette disposition est déjà satisfaite par les textes en vigueur, ne nous paraît pas apporter les garanties suffisantes, dans la mesure où la circulaire du 25 janvier 2016, qui fixe les modalités de délivrance de

Par cet amendement, nous souhaitons au minimum que le Gouvernement nous apporte une clarification sur le droit en vigueur, notamment sur la portée de la circulaire de janvier 2016. La parole

Ils tendent à rétablir l'article 26 , supprimé en commission, qui réaffirmait le principe selon lequel l'autorisation de travail est accordée de droit aux mineurs non accompagnés s'agissant d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Or cette disposition est déjà prévue par le droit positif. L'article L. 5221-5 du code du travail précise, à son deuxième alinéa : « L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. » Ainsi, les mineurs isolés étrangers ne sont nullement exclus de cette disposition.

ajoute que ne peuvent y faire obstacle ni les conditions d'opposabilité de la situation de l'emploi, définies par l'article R. 5221-22 du code du travail, ni l'examen de la demande au regard

Malgré la démonstration juridique solide faite par le rapporteur, je me rangerai à l'avis du ministre. Certes, au terme d'un raisonnement juridique impeccable, le Conseil d'État arrive à conclure que l'interprétation du texte en vigueur aboutit à reconnaître une autorisation d'office de ces contrats d'apprentissage. Mais je crois vraiment que la rédaction que nous proposons au travers de ces amendements identiques rend le texte beaucoup plus lisible et permet justement de répondre

qui est contre

qui est contre

Le cas est moins fréquent, mais il arrive que certains mineurs non accompagnés veuillent suivre un cursus universitaire. Cet amendement vise donc à faciliter l'attribution de la carte de séjour temporaire mention « étudiant aux mineurs non accompagnés, dont la sensibilité les porte vers la poursuite d'études universitaires et à qui n'est attribué le titre temporaire de séjour qu'à la condition du suivi d'une formation professionnelle. L'amendement

Ces amendements tendent à ajouter un cas de délivrance de la carte de séjour mention « étudiant » aux mineurs non accompagnés pris en charge par l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans et qui poursuivent des études supérieures à leur majorité. Aujourd'hui, la situation de chacun de ces mineurs est régie par les dispositions de l'article L. 313-11 du qui prévoit que la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui est délivrée de plein droit, sous réserve que soient respectés trois critères : le caractère réel et sérieux du suivi de la formation ; la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine ; et l'avis de la de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La circulaire Valls laisse déjà une certaine souplesse en la matière, en permettant la délivrance de cartes de séjour « étudiant » dans des cas très spécifiques. Les amendements sont donc partiellement satisfaits.

Cet amendement a pour objet de rendre l'évaluation de minorité des jeunes migrants non accompagnés plus efficace pour les services chargés de l'effectuer et, surtout, de réduire le temps de l'évaluation.

Cela limiterait aussi la multiplication des évaluations pour un même mineur.

à Mme Élisabeth Doineau. En préambule, je souhaite préciser que cet amendement doit être apprécié comme étant une invitation à une plus grande collaboration entre le juge des enfants et le juge des tutelles. Je n'ai aucunement la prétention d'interférer sur les attributions des uns et des autres, mais je tenais à signaler cette difficulté particulière que nous avions également repérée. Lorsque l'évaluation de la minorité donne un résultat positif et que l'isolement du mineur est constaté, la tutelle doit être assurée par le conseil départemental. Mais plusieurs difficultés liées au problème de la dualité entre le juge des enfants et le juge des tutelles font obstacle à cette évidence. Ainsi, alors que la minorité et l'isolement sont évalués par le conseil départemental et, éventuellement, d'ailleurs, par le juge des enfants, le transfert de la tutelle, qui devrait directement en découler, ne peut être décidé que par le juge des tutelles. Un jeune peut alors se retrouver sans tutelle pendant plusieurs mois. C'est pourquoi cet amendement vise à prévoir l'attribution d'une tutelle sans délai aux mineurs non accompagnés.

Je ferai la même remarque qu'à l'instant. L'objet visé par cet amendement est sans lien avec le présent projet de loi. Il y est proposé des dispositions qui modifient le code civil et s'appliquent aussi bien aux étrangers qu'aux Français.